d'observation ? ... Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée,

La dégradation du marché locatif est en effet accentuée par l'absence d'encadrement généralisé des loyers dans les zones tendues, par un manque criant de logements à prix abordables, ainsi que par l'insuffisante solvabilité des ménages les plus modestes.

agglomérations en tension locative, cette augmentation est d'ores et déjà encadrée par décret, en application de l'article 18 de la loi de 1989. La règle est que la hausse ne peut excéder le montant du dernier loyer, sauf dans trois cas : lorsque le loyer n'a pas été révisé depuis plus d'un an, lorsque le loyer est manifestement sous-évalué et lorsque des travaux importants ont été réalisés.

les outre-mer. J'appelle votre attention sur le fait que le dispositif de ces deux amendements identiques ne permet pas d'atteindre cet objectif, puisque le décret envisagé ne s'applique bien entendu qu'à l'article 6 de ce projet de loi pour lequel cette précision n'est pas indispensable. D'ailleurs, si ces amendements étaient

Le logement constitue un besoin fondamental. Or notre droit ne fait qu'entretenir et favoriser la multipropriété, d'un côté, et l'inaccessibilité à la propriété des jeunes ménages modestes, de l'autre. L'indice de référence des loyers est sensible au prix de l'énergie, qui ne peut qu'augmenter au regard des investissements nécessaires pour répondre à la transition écologique et pour garantir notre souveraineté Le Gouvernement prétend, à travers l'article 6 de ce projet de loi, soutenir le pouvoir d'achat des locataires. Je pense qu'il n'en est rien. Le plafonnement à 3,5 % était bien trop élevé et surtout provisoire. On ne réglera pas ici et maintenant les dysfonctionnements du marché de l'immobilier, mais une réponse sur le long terme doit être apportée. Le présent amendement vise à prévenir de manière pérenne toute hausse incontrôlée des loyers en plafonnant la variation de l'indice de référence des loyers publiés par l'Insee à 3,5 %, sauf

Concrètement, cela vise à interdire aux bailleurs d'augmenter les loyers alors qu'ils ont effectué d'importants travaux d'amélioration du logement- mise aux normes de l'électricité, par exemple, ou création d'un ascenseur dans un immeuble collectif -et qui représentent au moins la moitié d'une année de loyers. Je crois qu'il n'est pas dans l'intérêt des locataires d'interdire ce type d'évolution. Ce ne sont pas des augmentations indues et ces investissements ne peuvent pas être réalisés à fonds perdu par les bailleurs. La commission

et ceux de la métropole pour ce qui concerne les montants forfaitaires liés aux charges, ainsi que pour la prise en compte du nombre de personnes à charge. Si je comprends bien l'intention, il me paraît difficile de modifier ces critères de calcul sans réexaminer ceux qui sont propres aux outre-mer, comme la quotité d'effort personnel ou les loyers plafonds. Au demeurant, cette préoccupation me paraît partiellement prise en compte par l'article 22, visant à prévoir que le Gouvernement remette au Parlement un rapport portant sur l'évolution des zonages et les modalités de calcul des aides au logement, y compris outre-mer. La commission

des niveaux élevés des loyers et des prix d'acquisition des logements anciens, ou encore du nombre élevé des demandes de logement par rapport au nombre d'emménagements annuels dans le parc locatif social -, un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de concertation, fixe annuellement le montant maximal des prix d'acquisition foncière et immobilière, par mètre carré. Ce mécanisme, existant déjà pour les loyers, est étendu aux transactions immobilières, afin de donner un coup d'arrêt à la hausse exponentielle du niveau des transactions et à la spéculation.

Les APL doivent retrouver leur pouvoir solvabilisateur au profit des ménages aux revenus les plus modestes. Tel est l'objet de cet amendement, qui pour contourner les fourches caudines de la recevabilité financière

d'euros d'économies cumulées sur les APL par le Gouvernement au cours des cinq dernières années. Cette hausse ne doit pas non plus faire oublier que le forfait de charges ne couvre plus que 40 % des dépenses réelles, ou que le loyer plafond, qui sert au calcul des APL

ce débat politique. Je vous rappelle que le Sénat a voté, le 4 juin 2020, la proposition de loi de Cécile Cukierman, qui visait notamment à supprimer le mois de carence au détriment des bénéficiaires des APL et à procéder à une revalorisation. Cette proposition a été de nouveau transmise à l'Assemblée nationale par le président Larcher après les élections législatives, et je ne peux que vous inciter à demander à votre groupe de la faire inscrire à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Enfin, par votre amendement, vous posez la question de la stratégie que nous devons adopter pour soutenir le logement au bénéfice des moins favorisés. Faut-il agir fortement à travers des aides personnelles ou à travers les aides à la pierre pour que chacun ait accès à un logement abordable correspondant à ses besoins ?

M. Daniel Salmon. Par cet amendement, nous voulons faire appliquer les sanctions en cas de non-respect de l'encadrement des loyers, en systématisant les amendes prononcées par le préfet, de sorte que les propriétaires commettant une infraction courent un risque accru d'être sanctionnés. Alors que sévit une pénurie de logements, nous constatons de trop nombreux abus. Tout un chacun le rappelle, le prix des loyers ne cesse de grever les budgets des ménages, en augmentant les dépenses contraintes.

Une dizaine d'amendes auraient été prononcées. À Lille, où une dizaine de signalements auraient été effectués, le préfet a récemment prononcé une amende de 9 000 euros contre une société civile immobilière, pour un dépassement de loyer de 100 euros par mois. Il s'agit donc déjà d'une forte sanction.

que le locataire garde la possibilité de saisir le juge pour obtenir la diminution de son loyer. Je ne pense donc pas que l'augmentation du montant des amendes soit le coeur du problème. Il faudrait plutôt voir comment bien informer les locataires pour leur permettre de faire des signalements, et comment augmenter les contrôles de telle sorte que les organes de conciliation soient utilisés

évoluent donc pour une large part en dehors des mécanismes de marché. Si cette évolution bénéficie aux locataires, elle pénalise à due concurrence les propriétaires.

de référence fixé par le préfet tienne compte de l'inflation. Or l'inflation est d'ores et déjà prise en compte, puisque le loyer de référence est égal au loyer médian, lui-même calculé à partir des constats de l'observatoire local des loyers, selon les catégories de logement et les secteurs géographiques.

leur augmentation. Concrètement, il conduirait à imposer un loyer plus faible que les loyers actuels, et porterait une grave atteinte à deux principes constitutionnels régissant la location dans le parc privé : le droit de propriété et la liberté contractuelle.

est à Mme Cathy Apourceau-Poly. Dans la même logique, et toujours en lien avec la proposition de loi déposée par notre groupe, le présent amendement tend à faire baisser le niveau

Le Conseil constitutionnel s'est ainsi opposé au dispositif prévoyant que le montant du loyer de référence majoré et celui du loyer de référence minoré seraient fixés, non pas respectivement à +20 % et-30 % du loyer de référence, mais à l'intérieur de ces limites.

est à Mme Cathy Apourceau-Poly. Cet amendement vise à définir le complément de loyer. Depuis la loi ALUR, ce complément a fait l'objet d'échanges nourris et de jurisprudences qui viennent pallier une définition imprécise tant pour les propriétaires que pour les locataires. Dans certains territoires, les commissions départementales de conciliation signalent une augmentation des saisines relatives à la contestation du complément de loyer, ce dernier pouvant être utilisé par les propriétaires pour atteindre un niveau de loyer supérieur à celui permis dans le cadre du dispositif d'encadrement des loyers, hors charges, tout en paraissant respecter le loyer de référence majoré. Dans ce contexte, il est proposé de compléter la définition en s'inspirant d'exemples rencontrés sur le terrain. L'existence d'équipements ou de matériaux luxueux, qu'il

La précision de la définition du complément de loyer permettra également d'accompagner les propriétaires de bonne foi ainsi que les locataires dans l'exercice de leurs droits. Les relations entre propriétaires et locataires sur ce sujet s'en trouveront apaisées. Quel

sur la loi ALUR. Le Conseil a déclaré contraires à la Constitution les dispositions qui réservaient la possibilité d'un complément de loyer à « des caractéristiques de localisation ou de confort exceptionnels

insalubres. Dans certains cas, les situations que vous recensez sont imprécises, et ne renvoient à aucune référence juridique connue. Dans d'autres cas, l'excès de précision nuira aux locataires, empêchant le juge de sanctionner les propriétaires indélicats.

Quel est l'avis du Gouvernement ? Dans le cadre de l'expérimentation relative à l'encadrement des loyers, un complément de loyer peut être justifié par les caractéristiques de localisation ou bien de confort d'un logement, dans des conditions qui sont déjà précisées.

dans la mesure où cette interdiction de location rend superflue la question du complément de loyer. Cependant, si ces situations existent, elles sont inacceptables : votre amendement donnera un moyen d'action supplémentaire pour lutter contre les propriétaires. Pour

Il serait contre-productif de ne pas prendre cette décision, quand, en parallèle, votre gouvernement lui-même développe des dispositifs comme Action coeur de ville ou Petites Villes de demain.

la variation maximale de l'indice des loyers commerciaux (ILC), pour les petites et moyennes entreprises, pour les commerces qui font la vitalité de nos communes, de nos bourgs et de nos villages. Le

Cet amendement, proposé par M. Marseille, vise à plafonner à 3,5 % l'indexation des loyers commerciaux applicable aux commerçants, à l'instar du dispositif prévu pour les locaux d'habitation des particuliers à l'article 6. particuliers à l'article 6. L'ILC, sur lequel est assise l'indexation automatique des loyers des magasins, est calculé sur la base de l'inflation, à hauteur de 75 %, et de l'évolution du coût de la construction, à hauteur de 25 %.

il est proposé, par cet amendement, de le limiter aux plus petites entreprises. Afin de déterminer l'éligibilité au plafonnement, il est proposé de reprendre les critères d'accessibilité préalablement définis lors de la crise de 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.

et c'est certainement le plus important, le ministère a lancé des négociations entre bailleurs et locataires afin de tenir compte de la situation actuelle, fortement inflationniste. Ces négociations ont, semble-t-il, débouché sur un nouvel accord entre les parties, qui consiste à limiter,

d'une telle limitation aux PME, car il n'y aurait pas vraiment de sens à intervenir sur les loyers payés par de grandes enseignes, pour lesquelles le rapport de force est plus équilibré vis-à-vis des bailleurs. La commission émet donc un avis favorable

à tous les acteurs. Je tiens, ici, à saluer le sens de la responsabilité dont a fait preuve l'ensemble des parties prenantes, pendant ces concertations que nous avons menées tambour battant depuis jeudi dernier et j'ai le plaisir de vous annoncer que nous sommes parvenus à un « accord de place » sur ce sujet important. Je tiens à saluer la mobilisation et la détermination des parlementaires, et notamment de M. Lemoyne, pour trouver, à nos côtés, un compromis sur le sujet.

avec les représentants des commerces et avec les parlementaires ont confirmé cette intention : nous ne remettons pas en question la réforme structurelle du calcul de l'ILC. Nous avons, tous ensemble, trouvé une solution pour parer à l'urgence de la situation. Dans cet esprit, les concertations ont permis à l'ensemble des parties prenantes d'obtenir un accord de place, visant à répondre au contexte inflationniste. L'amendement défendu par Jean-Baptiste Lemoyne est le reflet de cet accord, qui consiste à plafonner temporairement à 3,5 % l'ILC pour les petites et moyennes entreprises,

0,3 point de plus, ce n'est pas anodin ! Madame la présidente de la commission des affaires économiques, je regrette que le seul amendement

parfois pendant plusieurs jours. Actuellement, il revient aux abonnés de faire les démarches pour obtenir un remboursement, alors même qu'ils ne sont pas à l'origine du dysfonctionnement. Celles-ci peuvent être longues, compliquées, comme les démarches peuvent parfois l'être. En conséquence, il semblerait nécessaire, dans ce cas précis, de rendre l'indemnisation

Mon amendement à cet article n'ayant pas été jugé recevable, je souhaitais évoquer cette mesure de bon sens. Je suis saisie

libellé : La parole est à Mme Sabine Drexler. Les entreprises proposent souvent à leurs clients un contrat avec une période d'essai gratuite, et lorsque celle-ci s'arrête, l'abonnement continue d'être prélevé automatiquement. Le client, n'ayant pas eu le temps de le résilier ou n'ayant pas reçu le message indiquant la fin de la période d'essai, continue de régler l'abonnement. La souscription ne doit pas être automatique et l'absence de réaction du consommateur ne vaut pas accord : il faut ainsi un accord exprès et renouvelé de sa part.

vise à permettre au consommateur de résilier facilement un contrat conclu par voie électronique. La localisation des entreprises ne doit pas constituer un obstacle à l'application

d'inscrire la généralisation de cette obligation dans la loi, afin de lever toute ambiguïté de lecture et d'éviter toute erreur d'interprétation. Par cet amendement, nous entendons préciser que le consommateur pourra résilier son contrat par voie électronique, que l'entreprise soit basée en France ou à l'étranger.

Par ailleurs, cet amendement crée un effet de bord important. En effet, si le consommateur n'a pas confirmé son souhait de continuer au-delà de la période gratuite, par exemple parce qu'il n'a pas noté à quel moment celle-ci prend fin, son contrat sera résilié alors même qu'il souhaitait certainement qu'il se poursuive.

de l'amendement n° 264 rectifié, il ne paraît plus nécessaire de repousser de six mois la date d'entrée en vigueur de l'article, lequel, je le rappelle, s'appliquera aux opérateurs qui savent déjà conclure des contrats par voie électronique. Les développements informatiques pourront donc être réalisés en six mois,

que les services de mon ministère sont prêts à examiner de très près cette question du remboursement en cas de dysfonctionnement de la ligne du fait de l'opérateur. Je suis à votre disposition pour que nous en parlions ensemble rapidement. Vous soulevez là un point

d'agir effectivement sur son pouvoir d'achat et de choisir un mode de consommation plus vertueux. L'amendement

Or, si les frais de résiliation de deuxième année disparaissent, il peut être légitimement entendu que le prix de l'équipement ou de l'abonnement va augmenter, la formule de calcul s'en trouvant profondément modifiée.

nous avons prévu que, pour de telles offres, des frais de résiliation pourront toujours être appliqués, mais sans dépasser le plafond de 25 % des sommes encore dues. Cela permettra d'éviter une hausse certaine du prix des téléphones et des abonnements tout en laissant la possibilité aux opérateurs

de ne pas appliquer la suppression de ladite règle aux contrats de communications électroniques couplant une offre de services avec l'acquisition d'un équipement terminal subventionné. Le rapporteur pour avis l'a également rappelé, le Sénat, en commission,

les contrats d'équipement et les forfaits. Cela s'appelle de la transparence ! Tel n'est pas le cas de tous les opérateurs, monsieur Chaize, et vous les connaissez très bien. La parole est à M. Victorin Lurel, pour explication de vote.

Pour exercer son droit de rétractation, le consommateur doit informer le professionnel de sa décision de se rétracter par l'envoi, avant l'expiration d'un délai de quatorze jours, du formulaire de rétractation ou de toute autre déclaration exprimant cette volonté. Ces exigences ne doivent pas être l'occasion pour les professionnels de maintenir des contrats et d'empêcher leur annulation par les consommateurs. Dans sa rédaction actuelle, l'article L. du code de la consommation permet déjà au consommateur d'exercer son droit de rétractation en ligne, que le contrat ait été conclu par voie électronique ou non. Cet amendement tend à offrir un cadre précis et facilité à l'exercice du droit de rétractation par voie électronique. Dès lors, et au même titre que pour la résiliation, il convient de mettre à disposition des consommateurs un accès électronique facilité pour cette rétractation.

ces contrats extrêmement bien ficelés, sans qu'il lui en soit donné copie. Ces sociétés utilisent ensuite les relevés d'identité bancaire remis par le client à l'occasion de cette opération pour prélever régulièrement de petites sommes qui n'attirent pas forcément l'attention. Les nombreuses réclamations portées à la connaissance des autorités et des associations de consommateurs font apparaître que ces remises et cadeaux sont des leurres. De même, les réclamations montrent montrent également que le consommateur est confronté, de la part de ces sociétés, à des montages et qu'il est parfois extrêmement difficile de joindre l'opérateur en question. Certes, et conformément à la loi Chatel, les sociétés d'assurance sont tenues d'informer avant terme le consommateur de la date d'échéance du contrat avant qu'il ne soit reconduit ; dans les faits, ces sociétés ne le font pas, et les réclamations sont extrêmement nombreuses. C'est la raison pour laquelle je vous propose de modifier l'article L. 113-15-1 du code

à tout moment les contrats de services de télévision et de vidéo à la demande. Cette disposition me semble disproportionnée. Premièrement, le code de la consommation, dans sa version actuelle, assure déjà un niveau élevé de protection du consommateur. Deuxièmement, il y aurait un risque d'incompatibilité avec le droit communautaire, le législateur européen ayant déjà écarté une telle disposition en 2019. Troisièmement, une telle mesure, en modifiant le modèle économique des acteurs, pourrait conduire à une augmentation du coût des offres de télévision, contribuant ainsi à une réduction du pouvoir d'achat. La parole est à M.

adopté en commission sont presque des exceptions. Ces dernières années, nous avons largement facilité le droit de résiliation de nombre de contrats, afin d'éviter que les consommateurs soient captifs

Je rappellerai quelques éléments essentiels. Tout d'abord, nous n'avons pas permis la résiliation à tout moment dès la conclusion du contrat. Ce n'est qu'après la première reconduction du contrat que le client bénéficiera de ce droit.

Il prévoit ainsi de renvoyer leur définition objective à un décret pris en Conseil d'État, afin, d'une part, de protéger davantage les consommateurs, et, d'autre part, de répondre à l'impératif de sécurisation juridique face aux écueils de la nouvelle disposition adoptée en commission.

comprenant une clause de reconduction tacite. Il vise ainsi à préciser que la résiliation à tout moment de ces abonnements est possible lorsque le consommateur déménage ou que son foyer fiscal évolue.

concernant les contrats de fourniture de contenus et services numériques, la directive européenne de 2019 a déjà tranché la question qui était en débat. Le législateur européen n'a pas souhaité interdire la tacite reconduction des contrats de fourniture de contenus numériques. En outre, je pose la question : pourquoi créer un régime spécial parmi les contrats prévoyant une clause de reconduction tacite pour les seuls contrats de fourniture de services de télévision ?

rectifié , rien ne dit quand le décret prévu sera pris, ce qui signifie que l'article pourrait rester inapplicable pendant des années. Par ailleurs, il serait étrange de préciser que, pour ces quelques contrats audiovisuels, le consommateur doit prouver qu'il a des motifs légitimes de vouloir résilier alors qu'il est libre de faire ce qu'il veut pour de nombreux autres contrats. Si vous souhaitez résilier votre abonnement à un service de vidéo à la demande ou à une chaîne de télévision, il n'y a pas à montrer patte blanche auprès de l'entreprise

le marché est suffisamment mature, et le modèle économique des opérateurs ne s'en trouverait pas modifié. En outre, nous ne revenons pas sur le principe de la tacite reconduction. Nous souhaitons simplement que les clients ne soient plus captifs de leur opérateur. S'ils souhaitent résilier une chaîne de télévision ou un service de vidéos à la demande, il me semble normal, à titre personnel, qu'ils puissent le faire sans attendre huit ou neuf mois.

trouve une réponse consensuelle et opérationnelle avec cet amendement. Celui-ci prévoit en effet que tous les contrats d'assurance, quels qu'ils soient ou quelle que soit la façon dont ils ont été conclus, sont résiliables par voie électronique, en quelques clics. Toutefois, pour ne pas pénaliser les petits acteurs,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

prévu par le texte initial du Gouvernement, soit le 1février 2023. En effet, selon l'étude d'impact, la mesure proposée ne constitue pas une contrainte ou une charge excessive et ne nécessite pas d'investissements importants de la part des professionnels du secteur,

agressive, dès lors que cette pratique est suivie de la conclusion d'un contrat, ce qui constitue une circonstance aggravante. Par ailleurs, pour ces délits, la peine d'emprisonnement est portée à sept ans lorsqu'ils sont commis en bande organisée. La peine d'emprisonnement est également portée à trois ans pour le délit de tromperie, qui, pour être constaté, suppose nécessairement la conclusion d'un contrat. Toutefois, nous regrettons que l'article 9 ne fasse pas suffisamment évoluer les amendes, qui sont plus effectives, donc plus dissuasives,

C'est là que réside le nerf de la guerre qui doit être menée contre les pratiques trompeuses, lesquelles portent atteinte au pouvoir d'achat, à la santé des consommateurs et à l'environnement.

également à supprimer l'alourdissement des sanctions dans le cas où ces pratiques seraient commises en bande organisée. Il me semble utile de nous assurer que les sanctions sont réellement dissuasives pour lutter contre les pratiques trompeuses. trompeuses. Ces dernières, ne l'oublions pas, ont un impact important à la fois sur la santé, sur l'environnement et, bien entendu, sur le pouvoir d'achat des consommateurs puisqu'elles les conduisent à engager des dépenses qu'ils n'auraient pas faites si on ne les avait pas trompés. Mme la ministre nous donnera peut-être des chiffres sur le montant de ces dommages.

C'est un vrai problème, car cela revient à traiter ces pratiques dommageables comme celles des dossiers sans grande importance. Surtout, je souhaite que la circonstance de bande organisée ne permette pas d'octroyer de nouveaux pouvoirs à la DGCCRF. Contrairement à ce que les acteurs du démarchage à domicile craignent, direction fera son enquête. Comme avant, elle transmettra les éléments au procureur, qui choisira ensuite, ou non, de placer une personne en garde à vue ou de déclencher des poursuites. À tout moment, si le juge considère qu'il ne s'agit pas d'une bande organisée, la qualification tombe. Cet article 9 tend donc à élargir non pas les pouvoirs de la DGCCRF, mais ceux de l'autorité judiciaire. Je me permets de signaler également que cet article vise à alourdir les peines de prison uniquement pour les cas où il y a eu conclusion d'un contrat. Cela ne concernera donc pas toutes les pratiques, mais uniquement les plus préjudiciables aux consommateurs- nous voyons tous très bien à quel type de pratiques je fais allusion. Je précise en outre que, compte tenu des règles de recevabilité, les amendements visant à interdire le démarchage téléphonique pour le compte personnel

à tromper les consommateurs. En revanche, il me semblerait utile que le Gouvernement explique plus clairement au Parlement la raison pour laquelle il demande l'adoption de ces mesures, qui n'entraient pas dans le champ des discussions menées autour de l'ordonnance prise récemment sur le même thème. La commission s'en remet donc à la sagesse du Sénat sur l'amendement n°

entre le premier semestre 2021 et le premier semestre 2022 ! De tels chiffres démontrent, s'il le fallait, qu'il est nécessaire de légiférer pour renforcer

Au regard de l'étude d'impact, il est apparu que l'autorité judiciaire retenait souvent la qualification d'« escroquerie » devant de telles pratiques commerciales déloyales. En 2020, plus de 16 000 escroqueries et abus de confiance ont donné lieu à des condamnations. Il convient d'affermir la peine applicable à ce délit en prévoyant une amende plus lourde, et ce afin de donner au juge une plus grande latitude de jugement

Le débat est en réalité plus large : les pouvoirs publics ne manquent pas d'outils financiers pour sanctionner ces pratiques, qu'on les appelle « pratiques commerciales trompeuses » ou « escroquerie ». En revanche, il faut maintenant faire un usage

nos importations sont réalisées par voie maritime, et nous sommes également tributaires de la situation oligopolistique qui voit trois compagnies se partager le transport de fret vers Wallis-et-Futuna. Le fret maritime a été multiplié par deux et le dispositif d'aide au fret institué par le décret n° 2017-1476 du 16 octobre 2017 est pour ainsi dire inopérant, car les activités bénéficiaires visées par l'arrêté préfectoral n° 2022-159 sont, sur place, Cette aide, qui peut aller jusqu'à 55 % des dépenses éligibles, ne s'applique pas non plus au transport de marchandises entre nos deux îles, Wallis et Futuna, à peine distantes de 200 Les fluctuations des cours mondiaux du pétrole affectent également l'évolution des prix ; ainsi nous retrouvons-nous aujourd'hui à subir une hausse du coût de l'énergie de plus de 7 %.

De plus, 90 % des banques n'informent tout simplement pas leurs clients de ce droit sur leur plaquette tarifaire. Un décret de juillet 2009 permet certes au client d'exiger le remboursement des frais perçus en cas de nouvelle tentative de prélèvement après un premier rejet,

marque automatique » des prélèvements infructueux, qui permet désormais aux établissements bancaires d'identifier facilement la répétition d'une même facturation. Cet amendement a donc pour objet d'imposer à ces établissements le remboursement des sommes indûment perçues.

consommation. L'article L. 612-39 du code monétaire et financier répertorie les sanctions pécuniaires que la commission des sanctions de l'ACPR peut prononcer

dispositions, cette nouvelle sanction qui, vous l'avez compris, ferait concurrence au cadre actuel, ou pourrait être interprétée comme telle, les établissements concernés verraient la sanction qu'ils encourent amoindrie. Cette sanction se limiterait en effet à imposer un remboursement des préjudices subis par les clients, alors que les sanctions actuellement prévues dans le code monétaire et financier peuvent être bien plus importantes- c'est pourquoi le Gouvernement a déposé cet amendement de suppression. Je comprends parfaitement

Or, l'an dernier, à l'occasion de l'examen de la loi Climat et résilience, la réforme du code minier a été renvoyée à des ordonnances, tandis que les responsabilités ont été transférées aux acteurs locaux. acteurs locaux. Conséquence directe aujourd'hui, les concessionnaires qui gèrent les anciens puits de mine, comme Gazonor chez nous, sont bloqués : l'écrasante responsabilité qui est devenue la leur les empêche de travailler convenablement. convenablement. Les projets de captage du gaz de houille, ou gaz de mine, ont été repoussés. Or ce gaz remonte déjà naturellement, et il est relâché dans l'atmosphère quand la pression devient trop forte. Nous pourrions amplifier l'expérience menée par endroits dans le Pas-de-Calais, à savoir injecter ce gaz gratuit dans les réseaux de chauffage urbain, mais cela suppose que l'on apporte des garanties aux acteurs locaux. J'avais déposé un amendement en ce sens, mais il a été déclaré

tandis qu'ici même nous allégeons les contraintes sur des procédés énergétiques plus discutables, comme l'importation de gaz de schiste ou de sables bitumineux. davantage une requête qu'une explication de vote : penchons-nous enfin sur la gestion de l'après-mine et engageons une refonte complète du code minier. Je demande, comme l'ont fait l'Association des communes minières, le conseil régional des Hauts-de-France et les deux départements du Nord et du Pas-de-Calais,

et j'en appelle à la poursuite d'une véritable planification énergétique. L'outil de stockage national se voit offrir la dimension stratégique et de résilience

Merci